ne peut présider notre séance, car il se rend actuellement en Côte d’Ivoire à l’invitation de la présidente du Sénat ivoirien, Mme Kandia Camara, dont il est l’invité d’honneur à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire du Sénat ivoirien et du colloque des Sénats africains qui doit aboutir à la création d’une association des Sénats d’Afrique. Mes chers collègues, je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau, j’appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole.

vous vous êtes longuement exprimé devant l’Assemblée nationale, puis devant le Sénat pour présenter votre déclaration de politique générale. À aucun moment lors de ces interventions, vous n’avez présenté précisément vos projets austéritaires, alors que vous aviez déjà en votre possession le projet de budget. Depuis se dessine la sanction lourde que vous allez imposer aux collectivités locales. Un effort de 5 milliards d’euros leur serait demandé, alors que nous connaissons tous

auxquelles s’ajouterait la baisse probable de 1 milliard d’euros des crédits du fonds vert. Cette ponction accrédite l’idée inacceptable répandue par MM. Le Maire et Cazenave que les collectivités seraient responsables de l’endettement. C’est honteux, alors qu’elles assument elles mêmes leur dette. Ce plan de casse du service public local est intolérable. Ce plan, c’est la mise à mal de l’investissement public local, alors même que les collectivités financent plus des deux tiers de l’investissement public de notre pays. Jusqu’à présent, les collectivités locales étaient souvent le dernier rempart contre les coups de boutoir du libéralisme, un bouclier contre la paupérisation et le repli sur soi de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, confirmez vous ce choix, votre choix, contre les collectivités, leurs élus, leur population, ce choix contre votre pays et ses territoires

D’abord, un fait : les dépenses des collectivités locales ont beaucoup augmenté depuis quelques années. Et je sais pourquoi. Je pense que cet argent a été bien utilisé, comme vous l’avez indiqué vous même, et que beaucoup de ces dépenses sont des dépenses subies ou contraintes en raison,

que nous devons gérer et qui crée une incertitude, un doute, tout autour de nous, en Europe, et aussi chez nous. Or nous avons un devoir de responsabilité, que j’assume, madame la présidente,

ans. Je ne mettrai donc jamais les collectivités locales en accusation. Jamais ! Je sais qu’elles gèrent, et cela au plus près des gens, des difficultés, des politiques publiques, des projets… Je n’ai pas oublié cette responsabilité. Pour autant, les mesures du projet de loi de finances que nous allons présenter demain préservent les principes auxquels je tiens. Ainsi, sous réserve de la discussion parlementaire, nous protégerons les collectivités les plus fragiles.

à travailler pour affiner cette orientation qui, je le crois, permettra de faire comprendre aux communes, malgré l’effort que nous devons faire ensemble – j’en ai parlé –, que nous souhaitons leur donner plus de libertés et leur faire davantage confiance. La

Monsieur le ministre, ce lundi 7 octobre, nous avons commémoré les terribles attaques terroristes qui ont endeuillé Israël l’an dernier. Aujourd’hui, alors que la France connaît une augmentation alarmante des actes antisémites, nous réaffirmons clairement notre solidarité avec Israël dans son aspiration à la sécurité et au retour des otages. Il nous faut également redire tout aussi clairement notre solidarité aux populations civiles qui souffrent et meurent tous les jours à Gaza ou au Liban. Le Hezbollah, qui gangrène le Liban, a entraîné le pays dans un conflit dont les Libanais ne veulent pas. Le Liban n’est pas le Hezbollah. Au Liban, pays frère de la France depuis près de mille ans, la situation humanitaire se dégrade de jour en jour. Plus de deux mille personnes ont déjà trouvé la mort. Des milliers de blessés affluent dans des hôpitaux saturés. Plus d’un million de personnes fuient le sud du pays. Des dizaines de milliers d’autres quittent la capitale bombardée. Monsieur le ministre, ce pays n’avait pas besoin d’une guerre. L’économie y était déjà à genoux. Il n’existe plus de classe moyenne, intégralement passée sous le seuil de pauvreté. Alors, la solidarité s’organise localement, mais elle ne pourra pas tenir longtemps. Les déplacés sont hébergés dans des écoles, des églises, des gymnases, bientôt dans des maisons vides. La population ne peut pas répondre seule aux besoins humanitaires immenses. Dans ce contexte alarmant, sur fond d’escalade dans toute la région, que peut la France, la tendre mère ?

Avant les opérations militaires israéliennes, la situation économique et sociale de ce pays était dramatique. Elle est aujourd’hui catastrophique. Vous l’avez rappelé, des milliers de morts, dont des enfants, des milliers de blessés, des centaines de milliers de déplacés ! Si rien n’est fait,

C’est la raison pour laquelle, sous l’autorité du Premier ministre, le Gouvernement agit. Il agit, d’abord, pour assurer la sécurité de nos ressortissants, celle de nos agents, mais aussi celle de nos militaires sur place mobilisés au sein de la Finul. Sophie Primas répondra tout à l’heure à une question à ce sujet.

de médicaments. Mais tout cela ne suffit pas ; c’est la raison pour laquelle je vous annonce que la France accueillera le 24 octobre une conférence internationale pour le soutien au Liban. Enfin, nous encourageons les responsables politiques libanais à prendre leurs responsabilités pour mettre le pays sur les rails, pour que le Liban conserve son unité et sa stabilité. Il faut que le Liban se dote d’un Président. C’est ce à quoi nous l’encourageons vivement. Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement mobilisé au service du Liban et au service de la paix.

et de la forêt. Madame la ministre, parlons dette écologique ! L’agriculture biologique connaît une crise sans précédent depuis trois ans. Les raisons en sont multiples : des engagements non tenus,

Tout semble fait pour freiner le développement de la bio. Les conséquences sont désastreuses : les agriculteurs bio sont de plus en plus nombreux à « déconvertir » leur ferme. Un immense gâchis d’argent public ! En 2023, les pertes économiques pour les agriculteurs bio ont été estimées entre 250 et 300 millions d’euros. Les surfaces en première année de conversion ont chuté ; la surface agricole utile (SAU) en bio stagne. Non, mes chers collègues, il n’y a pas deux modèles qui se valent. La bio a apporté les preuves scientifiques qu’elle est le label le plus abouti pour la santé et l’environnement. Ses externalités positives ne sont plus à prouver et on doit la payer pour cela. La bio n’est pas une niche, ni une option ; elle doit être le cap. Si l’État entend respecter l’objectif de 21 % de surfaces agricoles en bio d’ici à 2030, il n’y a plus de temps à perdre. Le fonds d’urgence de 105 millions d’euros mis en place en début d’année est largement insuffisant. Il est impératif de créer de nouveaux débouchés pour cette filière, impératif de poser les bases d’un financement équilibré de la bio dans la durée, comme le préconise le rapport de la Cour des comptes. Madame la ministre, vous engagez vous pour une politique ambitieuse, structurelle et de long terme pour sauver l’agriculture biologique ? La parole est à Mme la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Monsieur le sénateur

ont également été mises en place : un crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique à hauteur de 109 millions d’euros et plus de 50 millions d’euros pour l’écorégime. Sur la planification écologique, le budget du fonds Avenir Bio a été porté à 18 millions d’euros par an il est en hausse de 5 millions. Enfin, le budget de communication pour valoriser les productions bio a été porté à 5 millions d’euros par an pour soutenir une campagne de communication massive sur la consommation de ces produits.

agriculture. Elle fait vivre des agriculteurs et je veux vous dire très solennellement que je serai à leur côté par la politique que j’entends conduire en la matière. parole est à M. Daniel Salmon, pour la réplique.

l’effondrement de la biodiversité. Ce sont surtout énormément de coûts cachés dans notre système alimentaire. On estime ainsi à 19 milliards d’euros le coût sur la santé de l’alimentation actuelle. Faisons la vérité des prix ! Non, la bio n’est pas chère. Monsieur le Premier ministre, vous avez introduit

pays dans lequel vivent 180 000 de nos compatriotes. La France est attachée de manière indéfectible à la sécurité d’Israël. Et ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Lorsque le Hamas a perpétré contre Israël le pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, la France a sanctionné les responsables du Hamas.

Lorsque l’Iran menace la sécurité d’Israël en développant son programme nucléaire, c’est encore la France qui est en première ligne des efforts internationaux pour faire échec à ce programme. Nous considérons aujourd’hui que la force seule ne peut suffire à garantir la sécurité d’Israël et des Israéliens et que le recours à la force doit désormais céder la place au dialogue et à la diplomatie. C’est pourquoi la France, comme la plupart des pays dans le monde, appelle aujourd’hui au cessez le feu, à ce que la force cède la place à la diplomatie et au dialogue, à Gaza comme au Liban. Et lorsque l’on appelle à un cessez le feu, on ne peut pas en même temps fournir des armes offensives aux belligérants, quels qu’ils soient. La position de la France est constante sur ce sujet. C’est une question de cohérence.

Monsieur le ministre, j’apprends que la France a pris des sanctions contre les dirigeants du Hamas seulement après le 7 octobre ! J’ose espérer que cela a été fait avant, France, on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. Et je ne vois pas pourquoi il n’y aurait pas eu de sanction bien avant cette date. Monsieur le ministre, être amis, c’est se dire des vérités, c’est dire comment la France voit l’avenir de Gaza ou du Liban,

le monde… – que, depuis le 8 octobre de l’année dernière, le Hezbollah bombarde tous les jours les villes du nord d’Israël, et cela dans une indifférence quasi générale. C’est inacceptable ! Quel pays au monde accepterait que ses villes soient bombardées tous les jours et qu’on lui dise : « Surtout, ne réagissez pas. » Israël n’est pas un très grand pays, mais c’est un pays qui regarde beaucoup la France et les Israéliens se demandent : où est la France ? Est ce que la France sait encore où elle habite par rapport à nous ? Faites en sorte, monsieur le ministre, que les Israéliens retrouvent l’adresse de la France ! La parole est

Monsieur le Premier ministre, les blocages, les affrontements avec les forces de l’ordre ou encore les scènes de violences urbaines se propagent peu à peu à l’ensemble des outre mer. C’est le cas à Saint Laurent du Maroni en Guyane ou, ce lundi encore, en Martinique. Nous condamnons tous fermement ces actes de violence et appelons à un retour au calme. Pour autant, les causes de cette colère sont profondes en outre mer. À la Martinique, c’est une mobilisation citoyenne contre la vie chère, due à l’initiative d’une association, le RPPRAC (Rassemblement – ils sont 40 % plus élevés que dans l’Hexagone –, les ménages martiniquais sont littéralement asphyxiés, au mépris de la promesse républicaine d’égalité, de solidarité et de fraternité. Des propositions responsables, que je partage avec le président de la collectivité, Serge Letchimy, ont été faites à la suite de réunions de concertation avec le préfet et tous les acteurs concernés. Ces propositions pour faire baisser durablement les prix s’articulent autour de quatre axes majeurs. Premièrement, ramener à zéro la taxation de l’octroi de mer régional et de la TVA sur une liste de cinquante quatre produits de grande consommation. Deuxièmement, constituer un fonds, financé par l’État et les compagnies de transport maritime, afin de compenser les frais d’approche pour une liste de produits de première nécessité. renforcer la transparence et le contrôle des marges des distributeurs et des grossistes importateurs dans le respect du secret des affaires. accompagner l’autonomie alimentaire, en aidant la production agricole locale par plus de diversification et de structuration pour les filières existantes. Monsieur le Premier ministre, afin de valider ce protocole d’accord, des décisions doivent être prises en urgence par votre gouvernement. Aussi, ma question sera simple quand allez vous venir sur place ? Et quelles sont les mesures envisagées pour répondre au mécontentement légitime de la population martiniquaise ? La parole

les ont visées et que plus de trente policiers et gendarmes ont été blessés. Vous avez raison de dire que, partout sur le territoire de la République, l’ordre républicain doit être respecté, ce qui n’empêche pas de regarder en face les difficultés des Antilles, et de la Martinique en particulier.

Je ne pourrai y répondre dès cet après midi, mais sachez, monsieur le sénateur, qu’elles font partie des propositions actuellement étudiées et discutées avec la collectivité territoriale de Martinique ainsi que les acteurs économiques.

Je vous indique également que l’État s’engagera sur le renforcement des moyens de l’observatoire des prix, des marges et des revenus et, plus largement, sur l’objectif d’une meilleure transparence des mécanismes de formation des prix. C’est absolument essentiel

pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France est actuellement confrontée à une grave crise du logement. La chute des ventes du neuf – elles ont baissé de moitié au deuxième trimestre de cette année par rapport au premier trimestre de l’année dernière –, nous le prouve. Face à cette situation préoccupante, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a appelé les maires à « revitaliser la construction de logements ».

Par ailleurs, les recours contre les permis de construire se multiplient. Cette brochette de procédures crée de véritables blocages juridiques. Ces contestations retardent les chantiers de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et découragent parfois les investisseurs.

l’augmentation du volume de logements intermédiaires détenus par les organismes HLM ou la généralisation du permis d’aménager multi sites. Dans ce contexte, madame la ministre, quelles mesures concrètes le Gouvernement envisage t il de prendre

qu’il a décidé de faire un effort particulier sur la politique du logement, en prévoyant tout d’abord un ministère du logement de plein exercice, ce qui n’était pas arrivé depuis 2017.

Plusieurs mesures ont d’ores et déjà été annoncées dès le discours de politique générale. Elles sont, je crois, de nature à apporter de premières réponses. Le premier sujet est la relance de la primo accession. Le Premier ministre l’a dit avec précision, il importe de développer le prêt à taux zéro (PTZ) sur tout le territoire. Cet outil est ancien et a fait ses preuves, mais il a besoin d’être proposé en tout point du territoire, urbain comme non urbain,

Le deuxième sujet est la relance de l’investissement locatif. Pour loger étudiants, travailleurs, agents publics, plusieurs travaux, dus notamment à des parlementaires, ont déjà ouvert des pistes d’aménagement et j’amorcerai rapidement une série de consultations pour avancer sur ce sujet.

Parallèlement à son rôle diplomatique, la France se doit d’assurer la protection de nos compatriotes. Aujourd’hui, les 21 000 Français du Liban, en majorité franco libanais, sont extrêmement angoissés. Contrairement à d’autres pays qui ont décidé d’évacuer leurs ressortissants, nous n’avons pas, à ce stade, fait ce choix, estimant que les vols commerciaux permettaient aux Français qui le souhaitaient de partir. Or non seulement la situation est loin de s’améliorer, avec des bombardements fréquents sur la route de l’aéroport, mais, surtout, une partie importante de nos compatriotes manquent de ressources, que ce soit pour payer les billets d’avion, actuellement hors de prix, ou pour s’installer en France. Par ailleurs, ceux qui font ou feront le choix de rester seront confrontés à une perte d’activité. Pour les enfants, le suivi pédagogique peut difficilement être assuré. Un de nos lycées français, à savoir le lycée Abdel Kader, ne pourra pas, quoi qu’il arrive, rouvrir ses portes, puisqu’il est actuellement occupé par 3 000 déplacés ayant fui les premiers bombardements. Madame la ministre, beaucoup de questions se posent aujourd’hui, d’abord pour ceux qui veulent rentrer en France ou s’y installer pour la première fois : comment les aider à partir ? Comment les accueillir quand ils n’ont pas de famille ici ? Ensuite, pour les Français qui décident de rester : des aides sociales et de l’enveloppe des bourses scolaires ? Enfin, quel message adressez vous à l’ensemble de la communauté française du Liban,

et Républicain. Ma question s’adresse à M. le garde des sceaux. La guerre entre les gangs fait rage à Marseille. Un adolescent de 15 ans est abattu ; le gang adverse, qui a soif de vengeance, commandite un tueur à gages depuis une cellule de la prison de Luynes et, une fois encore, il y a un mort innocent, Nessim Ramdane, à qui je voudrais que nous rendions hommage. Ce mécanisme, nous l’avons décortiqué dans le rapport de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France. Le seul fait nouveau, aujourd’hui, c’est l’extrême jeunesse du tueur. Tueur à 14 ans, cela fait frémir Vous mesurez donc l’effroi des familles des victimes, le plus souvent des mères célibataires, dépassées par ce qui leur arrive et qui nous demandent de l’aide. L’effroi, aussi, des populations devant de tels actes de violence, qui empoisonnent leur vie quotidienne et qui leur donnent le sentiment que la République les a quittées.

le statut des repentis, en préparation depuis des mois ; la lutte contre le blanchiment, la corruption ; les conditions de détention des narcotrafiquants, car nos prisons sont des passoires, monsieur le garde des sceaux, et c’est depuis leur cellule que les narcos dirigent leur business. L’actualité vient une fois de plus de nous le démontrer, tout circule dans les prisons françaises : drogues, trafics en tout genre. Les surveillants disent saisir en moyenne quatre téléphones portables par cellule. Il est urgent d’agir Dès le mois de juillet, le rapporteur et le président de la commission d’enquête, Étienne Blanc et Jérôme Durain, ont déposé une proposition de loi. Elle a été retirée de l’ordre du jour à la demande du Gouvernement. Pourquoi ?

Il se développe et nous devons être à la hauteur en formulant un certain nombre de propositions dans les meilleurs délais. Des travaux avaient été entrepris par l’ancien gouvernement. Parallèlement, une

sur le centre pénitentiaire d’Aix Luynes. Il est évident que la poursuite d’activités criminelles depuis un centre de détention n’est pas admissible. Je vais poursuivre l’action déjà engagée par mon ministère pour lutter contre l’introduction de ces objets, qui sont tout à fait illicites en détention. La sécurisation des prisons, et par là même celle des surveillants et de nos concitoyens, est une priorité absolue de mon ministère. Je souhaite savoir

vendredi dernier, plusieurs maires du département des Pyrénées Orientales, dont je suis élue, ont appris que la gendarmerie nationale ne pourrait pas payer les loyers des biens immobiliers loués aux collectivités jusqu’à la fin de l’année. Elle n’en aurait tout simplement plus les moyens.

comment est il possible que, dans notre pays, l’État soit dans l’incapacité de payer ses loyers, qui plus est les loyers de nos casernes de gendarmerie ? Comment cela peut il se produire, alors que ces contrats de location ne sont pas apparus du jour au lendemain ni conclus dans l’urgence ? Ces dépenses immobilières figuraient, bien évidemment, dans la loi de finances pour 2024, alors comment expliquer à nos élus que les crédits correspondants n’existent pas ou plus ? J’ai bien conscience, monsieur le ministre, que vous n’êtes pas responsable de cette situation. Cependant, vous êtes aujourd’hui notre ministre de l’intérieur et c’est à vous d’en répondre. et c’est à vous d’en répondre. Quelles mesures prendrez vous pour permettre le paiement de ces loyers dans les meilleurs délais et pour que cette situation ne se reproduise plus à l’avenir ? Pouvez vous également nous assurer que le programme d’investissement pour la construction de nouvelles gendarmeries sera bien respecté ? La parole

considéré qu’il était absolument impossible de laisser les bailleurs sociaux, mais aussi les collectivités, sans réponse. J’ai donc pris la décision d’honorer la parole et les engagements de l’État. Nous allons faire deux parts

Celle ci exige que nous cessions les instrumentalisations politiciennes. Ce genre de situation ne devrait pas exister. Nous devons nous efforcer d’agir pour que cela ne se reproduise plus, car une telle défaillance n’est pas admissible dans un pays où l’État se doit de respecter ses engagements et de montrer l’exemple, notamment lorsque la sécurité des Français est en jeu. La parole

Nous n’avons eu de cesse, sur ces travées, d’avertir nos compatriotes sur les choix budgétaires qui ont été faits depuis sept ans. Des choix que nous avons toujours dénoncés comme iniques, et qui n’ont fait qu’organiser l’attrition des finances publiques, et ce avec le quitus permanent de la droite sénatoriale. Les résultats sont probants : déficit à la dérive, supérieur à 6 % du PIB, soit un écart de l’ordre de 50 milliards d’euros. Je dois reconnaître que le macronisme finissant a fait fort cette année. Plus fort que Lorsque vous nous alertez sur le niveau d’impéritie des gouvernements macronistes, je peine à trouver la cohérence qui est la vôtre, monsieur le Premier ministre, vous qui nommez comme directeur de cabinet celui là même qui officiait auprès de Bruno Le Maire voilà un mois. On ne change pas une équipe qui perd d’euros : voilà la somme qu’il vous faut trouver. Ce sont précisément les recettes fiscales détruites chaque année par le président Macron. Vous choisissez de récupérer deux tiers de cette somme en coupant dans les dépenses, comme votre prédécesseur : vous semblez plus à l’aise avec la purge des dépenses publiques qu’avec la potion fiscale des profiteurs de crise. Monsieur le Premier ministre, pour mettre fin à la crise, il faudrait commencer par ne pas l’aggraver. Et ce n’est pas en faisant porter le chapeau aux collectivités, comme l’a fait Bruno Le Maire, que vous y parviendrez. Les remontées de terrain à l’annonce des 5 milliards d’euros de coupes budgétaires sont édifiantes. Dois je vous rappeler que les collectivités territoriales sont déjà à l’os ! Ma question est simple : alors que la droite sénatoriale a toujours voté tous les budgets des gouvernements macronistes, comptez vous enfin changer de doctrine afin que les erreurs du passé ne se reproduisent pas ?

et je tiens le même discours devant les députés. Le redressement des comptes publics est néanmoins l’affaire de tous, et de toutes les administrations publiques.

L’État devra ainsi être le premier contributeur au redressement des finances publiques. Sur les 40 milliards d’euros d’économies qui seront faites pour redresser nos comptes publics et atteindre l’objectif de déficit public de 5 %, l’État prendra sa part à hauteur de 20 milliards d’euros

que les collectivités territoriales devront contribuer à hauteur de 5 milliards d’euros. Est ce que toutes les collectivités doivent contribuer de la même manière ? Non ! Est ce que l’hétérogénéité de la réalité des finances locales doit être prise en considération ? Oui

450 d’entre elles seront prioritairement mises à contribution. Nous le ferons notamment à travers un fonds de précaution avec une gouvernance des collectivités territoriales, auquel nous ajouterons certains mécanismes d’écrêtement de dynamique de TVA

Cozic, pour la réplique. Monsieur le ministre, l’effort reposera non pas sur l’État, mais sur les Français ! En ces temps difficiles, la justice fiscale, et je dirais même le pouvoir de vivre, ne sont pas des mots vains. Ils sont le préalable nécessaire à toute acceptation des efforts budgétaires que vous demanderez à tous les Français.

Monsieur le ministre, la semaine prochaine, vous serez en Nouvelle Calédonie. Vous avez fait le choix d’y effectuer votre premier déplacement dans les outre mer en tant que ministre. Je vous remercie de l’intérêt que vous manifestez ainsi à cette collectivité de la République qui traverse, depuis le 13 mai dernier, une crise politique, économique et sociale sans précédent, avec treize morts directement liés aux émeutes. Les Calédoniens entament leur sixième mois de couvre feu, après avoir connu douze jours d’état d’urgence. Je souhaite relayer auprès de vous, monsieur le ministre, les alertes de nombreux maires calédoniens qui sont aux prises avec de vrais dilemmes financiers et doivent arbitrer entre des dépenses qui sont toutes aussi essentielles les unes que les autres : transport scolaire, salaire des agents municipaux, cantine scolaire, subventions aux associations, et j’en passe. Comment reconstruire les édifices publics municipaux détruits, alors que les budgets de ces communes ne parviennent plus à assumer les charges de fonctionnement courant ? Les populations des quatre communes du Grand Nouméa sont tout particulièrement éprouvées, et plus encore nos 12 000 concitoyens du Mont Dore Sud, qui sont isolés depuis cinq mois. Après les annonces du Premier ministre dans son discours de politique générale, et dans la perspective de votre prochain déplacement sur place, pouvez vous, monsieur le ministre, indiquer à la Haute Assemblée les actions prioritaires que le Gouvernement entend engager au plus vite pour sortir la Nouvelle Calédonie de cette crise ?

Nous partageons, je crois, la volonté de porter au rang de priorité nationale notre souveraineté alimentaire. Le contexte difficile actuel suscite une immense attente du monde agricole, qui demande, vous le savez, une reprise rapide des débats sur la future loi d’orientation agricole. Aujourd’hui, c’est particulièrement de la filière volaille que je souhaite vous parler, parce qu’elle est emblématique de l’abandon, en France, de notre souveraineté alimentaire. La La Cour des comptes a publié en septembre dernier un rapport alarmant sur l’aviculture française. Elle nous dit deux choses. D’une part, la consommation de la viande de volaille progresse dans notre pays depuis une vingtaine d’années ; celle ci est en passe de devenir la viande préférée des Français.

instabilité sanitaire, avec l’influenza aviaire ; elle subit un déferlement de poulets ukrainiens, sans d’ailleurs que le consommateur puisse connaître l’origine de la viande présente dans les produits transformés la cible systématique d’associations qui, sous un vernis de défense de l’environnement ou, prétendument, du bien être animal, utilisent le contentieux juridique pour bloquer les projets de créations d’élevage. Madame la ministre, dans ce contexte, deux questions précises. Premièrement, comment allez vous agir concrètement vis à vis des importations déloyales et assurer la transparence quant à l’origine des volailles dans nos assiettes ? Deuxièmement, comment comptez vous défendre les exploitants contre les activistes anti élevage ? Comptez vous redéfinir le prétendu « intérêt à agir » à l’aune de la défense de notre souveraineté alimentaire ? La parole

de l’intrusion dans les bâtiments d’élevage leur marque de fabrique. Il faut être très clair : l’intrusion dans un lieu privé est condamnable.

tragédie qu’elle subit encore aujourd’hui dans une guerre qui n’est pas la sienne. Monsieur le ministre, vous le savez, les innombrables résolutions prises par la communauté internationale n’ont pas été efficaces. Bien au contraire, elles ont renforcé les intérêts de certaines factions, libanaises ou non, au détriment de ceux du Liban et du peuple libanais. On sait désormais à qui profite ce crime ! Nous nous interrogeons sur la réelle résurgence d’un plan ancien visant à la désintégration du Liban. Monsieur le ministre, vous l’avez dit, les liens entre la France et le Liban, pays plusieurs fois millénaire, sont séculaires et profonds. Cela a été démontré durant les siècles passés et l’est encore aujourd’hui ; je vous en remercie. Mais le peuple libanais attend avec espoir une action, une initiative internationale efficace qui mette fin à l’anarchie persistante et lui permette de reconstruire son pays afin qu’il retrouve la place qu’il mérite parmi les nations civilisées. Monsieur le ministre, comment la France entend elle aider la population libanaise ? Comment aidera t elle le Liban à retrouver durablement sa souveraineté territoriale et son indépendance politique ? à vous remercier pays que vous portez dans votre cœur, ce pays frère de la France – nous l’avons dit tout à l’heure – se trouve aujourd’hui au bord du gouffre, pour des raisons que vous avez très justement identifiées. La communauté internationale s’est mobilisée à plusieurs reprises pour définir le cadre qui permettrait d’assurer à la fois la sécurité d’Israël et la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban.

des prix de l’essence et du gaz, de la menace terroriste, ou de la question des migrations, tout se joue aujourd’hui, pour partie, au Proche Orient. C’est la raison pour laquelle, sous l’autorité du Premier ministre, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour porter un message de paix et pour œuvrer, par la voie diplomatique, afin que cesse le feu, afin que cessent les souffrances et afin que le Liban, dans son intégralité territoriale et sa souveraineté, retrouve sa vraie identité.

ses fonctions, votre prédécesseure a adressé un courrier au Premier ministre pour tirer la sonnette d’alarme sur le projet de budget du ministère. Elle jugeait la proposition de faire des économies sur les établissements d’enseignement supérieur « irréaliste et dangereuse ». Cette année, le nombre d’universités en déficit s’élève à soixante sur soixante quinze, soit le double de l’an passé. Après avoir subi les mesures Guerini, l’inflation, les surcoûts énergétiques et une annulation de crédits de près de 1 milliard d’euros en février dernier, nos universités sont à bout de souffle Les premières victimes de ces baisses de crédits, ce sont les étudiantes et les étudiants. On craint désormais des fermetures d’antennes locales, qui remettraient en cause l’accessibilité des études supérieures au plus grand nombre. Nos universités vont devoir retarder, voire annuler, des recrutements. Cette nouvelle détérioration du taux d’encadrement va remettre en cause la réussite de toutes et de tous. Pis, depuis la rentrée, on voit réapparaître d’interminables files d’attente d’étudiants et d’étudiantes pour l’aide alimentaire, sans compter les difficultés permanentes qu’ils rencontrent La baisse prévue des crédits remet en cause la revalorisation des bourses pour 2025, ainsi que l’acte II de la réforme des bourses sur critères sociaux. Cette précarité étudiante est une honte pour notre pays ! Monsieur le ministre, nos universités forment notre jeunesse et préparent l’avenir du pays. Saurez vous les défendre et empêcher qu’elles soient sacrifiées ?

quasi équivalent à celui que nous avons connu au cours des années précédentes. Vous le savez sans doute, puisque vous connaissez très bien ce secteur. On compte aujourd’hui 750 000 boursiers,

aux étudiants boursiers, ainsi qu’à ceux, auxquels vous faisiez référence, qui peuvent être en situation de précarité. Ce programme a offert, depuis un an, plus de 22 millions de repas. Encore une fois, l’effort de la Nation est réel.

Monsieur le ministre, je suis désolé, mais votre réponse n’est pas à la hauteur de la crise de la précarité étudiante. Je note d’ailleurs que vous n’avez pas repris ici une phrase que vous avez prononcée lors de la passation de pouvoirs : vous disiez alors que l’enseignement supérieur et la recherche, ce « n’est pas une dépense, c’est un investissement ». J’ai envie de vous dire : prouvez le en actes

qui ont signé une lettre envoyée récemment au Président de la République au sujet de l’avenir de la centrale Émile Huchet de Saint Avold. Pendant plusieurs semaines, les salariés de cette Ils sont inquiets, car le gouvernement précédent n’a pas apporté les réponses attendues. Ils sont inquiets, car, il y a un an, le Président de la République s’était engagé à convertir les centrales à charbon vers la biomasse d’ici à 2027 – ces promesses allaient dans le bon sens. Hélas, depuis, rien n’a avancé Mme Pannier Runacher s’était mobilisée pour la transition. Elle était venue sur le site et avait soutenu le projet hydrogène qui y était développé. Aujourd’hui, il y a urgence à agir Les contrats de travail d’une centaine d’emplois directs prennent fin en avril 2025, ce qui affecte les 150 sous traitants présents sur le site. Un projet de conversion à la biomasse ou au biogaz, qui permettrait de sortir définitivement du charbon en 2027, a été proposé par l’industriel exploitant du site. Ce projet garantit la sécurité d’approvisionnement et est conforme à la stratégie nationale bas carbone ; il vous Nous avons besoin d’une feuille de route claire pour la mise en œuvre des engagements pris par l’État. Dès lors, madame la ministre, ma question est simple : pouvez vous nous dire si les projets proposés seront soutenus, de manière à rassurer les salariés et les élus, à sauver des emplois et ainsi à tenir les engagements

clair : sortir des énergies fossiles et arrêter la production d’électricité à partir de charbon d’ici à 2027. Cette nécessité de décarbonation permet de lutter contre le changement climatique. Nous devons Nous devons désormais concilier cet objectif de décarbonation avec la recherche de solutions pour les sites concernés comme pour leurs salariés. Sachez, madame la sénatrice, que lorsqu’on s’est engagé, en tant qu’employé d’une entreprise, pour une activité, et que l’on apprend qu’il va falloir fermer, c’est difficile.

Agnès Pannier Runacher s’y était engagée en tant que ministre de la transition énergétique. Je reprends le flambeau, à ses côtés, pour que cette nécessaire transition écologique soit la plus juste possible et ne laisse personne sur le carreau.

d’autres projets encore sont à l’étude pour donner un avenir au site. L’État se tient aux côtés des salariés du site pour trouver, au plus vite, un projet créateur d’emplois, avec un modèle économique robuste et pérenne pour le territoire.

de vos promesses. Nous attendons maintenant des actes. Surtout, nous savons que trop d’emplois sont mis en danger par cette inertie. Madame la ministre, la transition écologique doit être une opportunité industrielle : ne laissez pas la Moselle à l’écart de celle ci

particulier dans les départements de l’est de la France, de la Meurthe et Moselle à la Haute Savoie. Au Luxembourg et en Suisse, les salaires sont deux à trois fois plus élevés qu’en France.

L’effet est double pour nos territoires. D’une part, ces anciens salariés restent souvent longtemps au chômage, alors même que bon nombre d’entreprises et de services publics frontaliers peinent à recruter. D’autre part, compte tenu de leur niveau de vie, ils contribuent au renchérissement du coût du logement.

Alors que l’État ponctionne, depuis 2023, une partie des excédents de l’Unédic, et à l’heure où Bercy cherche désespérément des recettes supplémentaires,

À Marseille, le 4 octobre, au bois de Boulogne, le 21 septembre, à Subles, le 29 septembre, Nessim, Philippine et Kylian avaient la vie devant eux, comme Thomas, Lola, Timothy, Laura, Mauranne et tant d’autres. Leur vie n’avait pas de prix et leur absence laisse une dette ineffaçable à l’égard de leur famille. Ils ont un point commun : leur mort était évitable. Ils sont les victimes de l’impunité organisée, du laxisme judiciaire, de l’immigration incontrôlée et du trafic de drogue trop souvent toléré. Or moins nous réglons ces problèmes sources, plus nous courons à la dépense sécuritaire. Il faut en urgence briser ce cercle vicieux de l’insécurité, d’abord et avant tout pour son prix humain, mais aussi pour son coût financier démentiel. les mafieux commanditent les assassinats depuis les prisons et appellent la police pour s’en vanter. Encore ce matin, le tristement célèbre cartel DZ Mafia – DZ veut dire Algérie – diffusait une allocution publique pour donner son point de vue sur la situation : l’humiliation est complète pour les institutions ! Les Français n’attendent pas un tournant d’austérité, mais un tournant d’autorité. Monsieur le Premier ministre, vous avez là un gisement de popularité et d’économie garanti. Mais pour cela, il faut assumer la rupture ! Ma question est donc simple : accepterez vous de lever le tabou du coût de l’insécurité en proposant à la Cour des comptes d’évaluer annuellement son montant exact ?

où peut on faire baisser la dépense publique sans abîmer les services publics de proximité dont bénéficient nos concitoyens ? D’abord, il nous faut savoir retirer les boucliers de protection que nous avons mis en place pendant les crises. L’argent public a été abondamment utilisé pour protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment face aux hausses des factures d’électricité. Nous devons aussi faire gagner en efficience la dépense publique.

au sein de cet hémicycle, pendant de longues semaines, mais nous devons aussi savoir assumer les priorités du Gouvernement : la sécurité de nos concitoyens est l’une

La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010 837 et de la loi n° 2010 838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable (39 voix pour, aucune voix contre) à la nomination de M. Jean Castex aux fonctions de président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. groupe Union Centriste, la discussion de la proposition de loi visant à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes, présentée par M. François Bonneau et plusieurs de ses collègues

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, la vie d’élu est d’abord un engagement personnel, pas toujours un engagement rationnel, au service de sa commune et du collectif pour un CDD qui sera renouvelé selon son choix ou celui des habitants.

Qui plus est, les élus des communes rurales font face à de plus en plus d’incivilités. Le constat est là : près de 10 000 élus ont démissionné depuis 2020, ce qui souligne la gravité de la situation. Dans nos territoires ruraux, la dynamique démographique et sociale évolue. Les petites communes, qui constituent l’essence même de notre tissu rural, sont confrontées à des défis de plus en plus complexes. L’un des problèmes auxquels elles font face est la difficulté à maintenir un conseil municipal complet et opérationnel atteindre le quorum indispensable pour tenir les réunions du conseil municipal se transforme parfois en obstacle récurrent. Avec un nombre de conseillers fixé sans réelle considération des réalités locales, il est courant de constater que des conseils municipaux peinent à réunir suffisamment de leurs membres pour pouvoir délibérer. Cette situation paralyse les décisions et compromet le bon fonctionnement de la commune.

Ces départs en cascade provoquent des situations d’instabilité, imposent la tenue d’élections partielles et plongent certaines communes dans d’infinies complications. Cette instabilité fragilise nos institutions locales. Par ailleurs, le processus électoral lui même pose problème. Constituer des listes électorales complètes se révèle un véritable casse tête. Dans de nombreuses communes, certains candidats se présentent uniquement pour compléter des listes, sans avoir le temps ni la volonté de s’engager dans la vie municipale. Lorsque la liste n’est pas complète, la commune risque de se retrouver sous tutelle préfectorale, une situation qui ne peut être tolérée dans une démocratie locale comme la nôtre. Au fil des ans, ce désintérêt se transforme en absentéisme lors des réunions, compromettant ainsi l’équilibre et l’efficacité du conseil municipal. Il faut souligner l’inadéquation entre le nombre de conseillers municipaux requis et la réalité démographique de nos communes rurales. Dans certaines d’entre elles, le conseil municipal représente jusqu’à 10 % de la population totale, tandis que, dans les grandes villes, ce pourcentage est infime. Ce décalage rend nécessaire une réévaluation des exigences en matière de représentation. Il est impératif de les rééquilibrer pour éviter des distorsions qui mettent en péril leur fonctionnement démocratique. En 2023, la France comptait 3 379 communes de moins de 100 habitants et 14 977 communes de 100 à 500 habitants. Si l’on s’en tient à l’état actuel du droit, cela représente 23 653 élus pour les communes de moins de 100 habitants et 164 747 élus pour celles comprises entre 100 et 500 habitants. Ces chiffres nous rappellent combien la France est majoritairement rurale et combien l’engagement citoyen est important pour nos villages. L’objet de ma proposition de loi visait initialement ces communes, qui sont les plus touchées par la difficulté de constituer une liste. Le texte dont nous discutons aujourd’hui vise donc à adapter le nombre de conseillers municipaux à la réalité des petites communes et s’inscrit dans le droit fil de la réforme du statut de l’élu pour mieux accompagner les représentants de nos communes.

villes de 2 500 à 3 499 habitants. Cette réduction permettra non seulement de faciliter la prise de décision, mais aussi d’assurer une gestion municipale plus efficiente et plus proche des besoins réels. Quand bien même un certain nombre de nos collègues voudraient que l’on donne toute latitude aux communes pour définir le nombre de leurs élus, une telle mesure se heurterait au Conseil constitutionnel et pourrait conduire à des disproportions importantes entre communes. Nous ne devons pas perdre de vue que nos communes rurales sont souvent les premières victimes des rigidités administratives. Cette situation est d’autant plus problématique que, si l’on exclut les résidents non permanents et les étudiants, le nombre de personnes éligibles se réduit drastiquement.

Il est également important de rassurer ceux qui craignent une diminution de l’influence des petites communes au sein des intercommunalités et du corps électoral des grands électeurs. La proposition de loi se limite à réduire le nombre de conseillers municipaux au sein des conseils, sans toucher à leur poids politique et à leur influence dans les instances intercommunales

supérieures. Mes chers collègues, cette proposition de loi s’inscrit dans une démarche de bon sens et de pragmatisme. Elle répond à un besoin de nos petites communes, qui doivent pouvoir fonctionner de manière plus fluide et plus efficace. En adaptant le nombre de conseillers municipaux à la réalité démographique et en simplifiant les exigences administratives, nous permettons à nos élus locaux de mieux gérer leurs dossiers et le quotidien de nos concitoyens. La mairie constitue bien souvent la porte d’entrée pour tout type de démarche, et c’est un service précieux.

je vous invite à soutenir cette proposition de loi, non seulement pour le bien de nos petites communes, mais aussi pour préserver et renforcer la vitalité de notre démocratie locale. Ensemble, faisons en sorte que nos communes puissent continuer à être des lieux de vie, de solidarité et d’engagement citoyen. La parole Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous sommes actuellement confrontés à une véritable crise des vocations à l’échelon local, régulièrement mise en lumière par les travaux du Sénat. Elle s’illustre notamment par l’accélération des démissions d’élus locaux en cours de mandat 1 787 maires, soit plus de 5 % des maires élus en 2020, avaient démissionné de leur mandat au début du mois d’octobre 2024, ainsi que 29 000 conseillers municipaux, soit 6 % d’entre eux. Des chiffres sans précédent également par la diminution du nombre de candidats aux élections locales. En 2020, après le dernier renouvellement général des conseils municipaux, 345 communes ne disposaient pas d’un conseil municipal complet contre 228 en 2014, soit une Cette situation a engendré de nombreuses difficultés de fonctionnement pour les conseils municipaux, particulièrement dans les communes rurales. Cela se traduit par le recrutement de conseillers municipaux moins motivés et moins investis dans leur mandat, un absentéisme plus élevé et des élections municipales complémentaires plus fréquentes. Cette crise s’explique principalement par la dégradation implacable des conditions d’exercice des mandats locaux, régulièrement dénoncée par le Sénat : hausse intolérable des violences contre les élus locaux, indemnités et garanties insuffisantes pour compenser leur engagement, complexification générale des affaires publiques locales, poids croissant des exigences citoyennes, manque d’autonomie financière et de reconnaissance. Ces obstacles entravent l’action concrète de terrain et concourent gravement au mouvement de désengagement observé. Pourtant, les élus locaux sont bien les garants de la préservation du lien social ; ils sont les sentinelles de la République. Nous avons besoin que ces femmes et ces hommes continuent de s’engager pour la vie de nos communes et de nos concitoyens. l’initiative du Sénat, des mesures fortes ont déjà été prises pour tenter d’entraver cette tendance inquiétante. Je pense notamment au statut de l’élu et à l’entrée en vigueur de la loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. J’en viens à la présente proposition de loi, déposée par notre collègue François Bonneau, dont je salue l’initiative et avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration. Je tiens également à remercier l’ensemble de mes collègues cosignataires du texte que j’ai moi même déposé sur ce sujet. Afin de combattre la crise des vocations dans la perspective des élections municipales de 2026 et de renforcer l’attractivité des mandats municipaux, l’article unique de la proposition de loi prévoyait initialement d’abaisser le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 500 habitants, plus précisément de sept à cinq dans celles de moins de 100 habitants et de L’objectif est de permettre aux communes rurales de constituer plus facilement leur conseil municipal, dans un contexte où le nombre de conseillers municipaux peut parfois excéder le nombre d’administrés disponibles pour un engagement citoyen.

alors que, pour la commune de Châteauroux, qui compte 43 000 habitants, l’effectif exigé représente 0,09 % de la population. là d’un écart considérable en termes de représentativité de la population municipale au sein du conseil municipal entre les petites communes et les villes moyennes. La commission des lois a donc accueilli favorablement cette initiative, qui, si elle ne résout pas les causes de la crise des vocations municipales, permettra aux communes rurales de constituer leur conseil municipal plus facilement.

d’abord, la commission a étendu la baisse du nombre de conseillers municipaux à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants, qui sont confrontées à des tensions grandissantes pour mobiliser suffisamment de candidats. Cette extension aura le mérite de favoriser la constitution des listes. Ensuite, la commission a souhaité modifier l’effectif des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants pour éviter une baisse trop brutale du nombre de conseillers municipaux dans ces communes et ne pas pénaliser celles qui réussissent à mobiliser suffisamment de candidats. L’effectif des conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants serait donc fixé à

ce qui leur laissera de la souplesse. Ainsi, les communes de moins de 100 habitants devront réunir sept conseillers municipaux, mais leur conseil municipal sera « réputé complet » ce qui permettra notamment d’élire un maire sans procéder préalablement à des élections complémentaires pour pourvoir les postes vacants. De même, les communes de 100 à 499 499 habitants devront réunir neuf conseillers municipaux, mais leur conseil municipal pourra être « réputé complet » avec sept conseillers municipaux. Qui plus est, la commission a apporté deux modifications pour garantir l’opérationnalité du dispositif et ainsi éviter tout effet de bord non souhaitable part, l’abaissement du nombre maximal de conseillers forains dans les communes de moins de 500 habitants, afin d’éviter que leurs conseils municipaux ne soient en quasi intégralité composés d’élus ne résidant pas dans la commune ; d’autre part, la garantie pour les communes concernées par la baisse du nombre de conseillers municipaux

Je tiens à insister sur un point : si ce texte constitue un progrès, il est urgent d’agir parallèlement pour résoudre les causes de la crise de la démocratie locale en enrayant enfin la dégradation des conditions d’exercice des mandats locaux.

le bénéfice de ces observations et sous réserve de l’adoption d’un amendement de coordination et de trois amendements identiques sur l’extension du principe du « réputé complet » pour les communes de 500 à 999 habitants, la commission des lois vous propose d’adopter cette proposition je vous remercie

le cœur de notre démocratie, le premier kilomètre d’une action publique efficace. Comme élus et comme citoyens, nous savons tous dans cet hémicycle à quel point l’engagement municipal est précieux, exigeant et ce qu’il représente dans nos vies.

retrouve ses concitoyens à la boulangerie ou dans la rue, prête toujours une attention bienveillante à tous et cherche à inventer des possibles pour améliorer le quotidien de chacun. Rendre ainsi service à ses concitoyens sur un territoire auquel on est attaché, en y consacrant tant d’énergie et de générosité, c’est la force, la vitalité, mais aussi l’honneur de notre République, l’illustration de ce que la délégation aux collectivités territoriales

Dans son discours de politique générale ici, au Sénat, le Premier ministre a clairement exprimé la haute idée qu’il se fait du rôle de nos collectivités locales dans la République. Il a appelé à bâtir un « nouveau contrat de responsabilités entre les collectivités

de mars 2023, 1 466 élections partielles se sont tenues du fait de l’incomplétude des conseils municipaux.

par l’adoption d’une proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, présentée par le sénateur François Bonneau et le groupe Union Centriste, dont je salue l’initiative, et signée par nombre d’entre vous, est la première pierre

apporte une réponse attendue aux difficultés des 18 000 communes de moins de 500 habitants dans la constitution de leur conseil municipal, en abaissant le nombre d’élus.

par votre chambre, à l’image de celle de Mme la rapporteure et du sénateur Éric Kerrouche. Je salue également tout particulièrement le travail utile auquel ont contribué votre rapporteure, Éric Kerrouche et Didier Rambaud et qui a conduit à l’adoption du rapport d’information sur l’efficacité du fonctionnement des conseils municipaux, le 3 octobre dernier, Ce travail collectif et transpartisan a élargi la réflexion sur le nombre de conseillers municipaux à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants, confrontées à des difficultés diverses de constitution d’assemblées municipales. Le Gouvernement partage la nécessité de traiter ce sujet en retenant un nombre adapté d’élus à la situation de chaque

Il nous semble nécessaire de veiller au respect des strates existantes, car chacune d’elles prévoit des droits et des devoirs pour les communes concernées : veillons à ne pas bouleverser ce qui ne pose pas véritablement problème Au vu des échanges avec les associations d’élus, il ne semble pas pertinent de modifier la loi pour les communes de plus de 3 500 habitants,

sur la représentation des communes de moins de 3 500 habitants au sein du collège électoral du Sénat, et c’est heureux ! Le Gouvernement est très attaché à la préservation de la représentation de toutes nos communes, en particulier des communes rurales, de la désignation de la Chambre haute. Aussi, nous n’approuverons pas les amendements dont l’adoption conduirait à une remise en cause de la place des plus petites communes dans le collège électoral des sénateurs. Il y va de la préservation de ce lien essentiel entre le Sénat et tous les territoires.

dans un esprit de dialogue, comme le souhaite le Premier ministre. Je connais la persévérance, l’obstination et la détermination du Sénat. Je sais que nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet. de revenir sur ce sujet. Monsieur le président, madame la ministre, chère Catherine Vautrin, madame la rapporteure, monsieur le sénateur Bonneau, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes tous très profondément attachés à l’engagement citoyen des élus locaux, parce que nous pensons que la commune est le fondement de la République, que les élus locaux en sont le cœur et que nous devons leur donner les moyens de réussir.

m’en réjouis, l’engagement du Premier ministre, du Gouvernement, et tout particulièrement de la ministre Catherine Vautrin, d’œuvrer ensemble, État et Parlement, pour élaborer des solutions concrètes et utiles pour notre démocratie. La parole

la République et la démocratie vivent dans nos territoires grâce à l’engagement des élus locaux, notamment des maires et des conseillers municipaux. J’ai le plaisir de saluer l’engagement de M. Pierre Colomb,

élus français. Mais force est de constater l’existence d’une crise de l’engagement local, notamment dans les plus petites communes de France. Selon les données du ministère de l’intérieur, lors des élections municipales de 2020, 106 communes n’avaient aucun candidat.

notamment dans les communes de moins de 500 habitants, nécessitant parfois l’organisation d’élections partielles. Plusieurs causes permettent de comprendre un tel contexte. On peut penser à la dégradation des conditions d’exercice des responsabilités locales, à la multiplication des violences et des menaces envers les élus, à l’inflation normative ou encore au manque de reconnaissance de leur engagement. Mais il faut également avoir en tête d’autres raisons constituer des listes complètes lors de chaque scrutin municipal, de réunir les quorums légaux, de respecter la parité. Toutes ces contraintes, certes justifiables, représentent néanmoins un véritable casse tête récurrent pour les élus et pour celles et ceux qui souhaitent le devenir.

La réduction du nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 500 habitants et de moins de 100 habitants est aujourd’hui nécessaire, comme elle l’était en 2013, lors de la précédente diminution. Et l’extension de cette diminution aux communes de moins de 3 500 habitants me semble également pertinente.

Je pense donc que ce texte, examiné sur l’initiative de notre collègue François Bonneau, apporte, grâce au travail réalisé en commission, une réponse adaptée, équilibrée et utile à la crise de l’engagement et bien plus adéquate que ce qui figurait dans la proposition de loi initiale.

la proposition de loi que nous examinons s’appuie sur un constat partagé et éprouvé par nombre d’entre nous : la crise de l’engagement public local. local. Cette crise est perceptible dans nos territoires, que ce soit dans les conseils municipaux, dans nos associations, auprès de nos aînés ou même dans nos entreprises. Or une société fragmentée est une société désarmée dans laquelle l’idéal républicain ne peut pas s’épanouir.

la proposition de loi constitue une tentative louable, elle ne nous empêchera pas de remettre sur la table des réflexions globales sur l’engagement public local, donc sur le statut de l’élu protecteur, ainsi que sur le scrutin de liste pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Les règles électorales doivent être claires ; elles fondent la confiance des Français dans leurs représentants. La proposition de loi initiale concernait les communes de moins de 500 habitants. Comme cela a été souligné, la commission a étendu

telles questions, légitimes, partagées et relayées par les maires eux mêmes, devraient nous conduire à prendre le temps de la concertation, faute de quoi nous risquerions d’adopter une norme difficile à comprendre. À une bonne et réelle question, soulevée aujourd’hui par le groupe Union Centriste, sachons ne pas apporter une réponse trop hâtive. Madame la ministre, chère Françoise Gatel, je sais que le Gouvernement est prêt à discuter, après consultation des concernés, d’une loi sur le statut de l’élu protecteur,

je tiens tout d’abord à féliciter l’auteur de cette proposition de loi, le sénateur François Bonneau, de son initiative tout à fait bienvenue. La question des effectifs des conseils municipaux est en effet souvent évoquée par les maires que je rencontre.

Le Sénat avait alors mis en garde contre une réduction du nombre d’élus locaux qui se ferait « automatiquement au détriment des territoires ruraux », et il n’avait finalement pas modifié les effectifs des conseils municipaux, contrairement à ce que proposait le gouvernement de l’époque. la vie locale et à la proximité de l’action publique a ouvert la possibilité de considérer comme étant complets les conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants et de moins de 500 habitants lorsqu’ils réunissent respectivement cinq et neuf membres, à défaut des sept et onze membres prévus par le code général des collectivités territoriales. La proposition de loi que nous examinons s’inscrit donc dans le prolongement de plusieurs initiatives législatives relatives aux conseils municipaux des petites communes.

J’ai souvent l’occasion d’évoquer avec les élus de l’Eure la question dont nous débattons aujourd’hui, et je constate que les avis sur le sujet sont partagés.

À cela s’ajoute la question du nombre d’adjoints, qui dépend directement du nombre de conseillers municipaux. En l’état, réduire le nombre de conseillers municipaux peut entraîner une diminution du nombre d’adjoints, qui n’est pas toujours souhaitée, tant s’en faut. Face à des attentes différentes, je pense donc qu’il est indispensable d’offrir de la souplesse aux élus. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement tendant à permettre aux communes de moins de 3 500 habitants de choisir le nombre de leurs conseillers municipaux avant leur renouvellement, dans une fourchette comprise entre ce que prévoient respectivement l’état actuel du droit et le texte de la commission. Très bien ! J’avais également déposé un amendement visant à garantir aux communes nouvelles le droit de conserver le même nombre d’adjoints à l’issue du deuxième renouvellement suivant leur création.

puis, dans sa version à enveloppe constante, au titre de l’article 45 de la Constitution. Je le regrette vivement, car il visait à répondre à une réelle préoccupation de bon nombre d’élus de communes nouvelles. Mes chers collègues, l’objectif du texte est majoritairement partagé par les territoires. Mais, encore une fois, une réduction imposée, rigide et uniforme du nombre de conseillers et d’adjoints créerait, de mon point de vue, des problèmes, et elle serait mal accueillie par les élus locaux, qui sont déjà soumis à rude épreuve. La parole

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour tenter de lutter contre un phénomène que nous connaissons bien et que nous combattons collectivement de manière constante : la crise de l’engagement local.

lors des élections sont – hélas ! – habituelles et devenues significatives lors du renouvellement de 2020. L’enquête confiée à l’institut CSA par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales au mois de montre que plus de la moitié des 500 élus interrogés dans les communes de moins 3 500 habitants ont rencontré des difficultés à réunir des candidatures aux élections municipales de 2020.

99 élus de communes de moins de 3 500 habitants avaient alors répondu. Un nombre important d’élus interrogés sont en effet favorables à une réduction du nombre de conseillers, au motif

Nombreux sont les élus locaux qui témoignent de l’abondance des tâches qui leur incombent et de leurs responsabilités. Mais comment faire toujours plus avec moins de moyens humains ? Par ailleurs, qu’en est il de l’enjeu de la représentativité ? Moins de conseillers, cela signifie moins de diversité au cours des débats, mais aussi moins de relais pour les habitants et leurs préoccupations. Nous retrouvons bien là la dichotomie dichotomie entre les communes comptant de 500 à 1 000 habitants et les communes de 2 000, 3 000, voire quasiment 3 500 habitants. Nous savons tous que les élus de nos communes, souvent bénévoles, sont fortement sollicités. Diminuer leur nombre risque donc de les pressurer davantage. Le texte initial prévoyait une réduction drastique pour les communes de moins de 500 habitants. Le travail en commission

la vie de la cité. Selon nous, l’engagement politique ne saurait se réduire à une carrière professionnelle. Voilà ce qui inspire nos propositions et nous permet de définir une vision claire des orientations nécessaires pour le bon fonctionnement de nos collectivités territoriales. Nous sommes tous à l’écoute de nos territoires ; nous connaissons la grande fatigue des élus au plus près des citoyens. Néanmoins, n’oublions pas que la France compte près d’un million de candidats sur les listes

Cela a des conséquences directes et rapides, en particulier sur les petites communes, qui peinent à obtenir ou à maintenir un nombre de conseillers municipaux suffisant pour agir. En ramenant le nombre

cela nous paraît d’ailleurs mieux adapté face aux problèmes de fonctionnement de nos institutions locales, au sein desquelles l’engagement devient trop compliqué. La rapporteure a aussi choisi d’étendre la réduction du nombre de conseillers municipaux aux communes comptant jusqu’à 3 499 habitants.

Monsieur le président, mesdames les ministres, madame la rapporteure, mes chers collègues,

a continué ses travaux sur l’efficacité du fonctionnement des conseils municipaux. Je tiens à remercier le sénateur François Bonneau, grâce à qui ce texte a été inscrit à l’agenda du Sénat alors que les élections municipales arrivent à grands pas. également Mme la rapporteure Nadine Bellurot pour la justesse de ses propos. Je rappellerai d’abord que les petites communes sont le cœur battant de notre démocratie locale, un espace où s’expriment pleinement les valeurs de la République et où se forge le lien de confiance entre les élus et les habitants. Et pourtant, elles sont particulièrement touchées

Ce texte est une réponse à un phénomène que nous connaissons bien : la difficulté croissante, pour les petites communes, de constituer des listes complètes lors des élections municipales. Dans le département dont je suis élu, l’Indre et Loire, nombre de communes

une action forte et adaptée. Par ailleurs, la réduction du nombre de conseillers municipaux n’est pas une décision publique anodine. Elle doit faire l’objet d’une analyse particulièrement fine et s’accompagner d’une nécessaire souplesse. Lors de l’examen du texte en commission, nous avons émis un avis réservé, considérant qu’une réduction permanente et uniforme des effectifs dans l’ensemble des différentes strates ne constituait pas toujours la réponse la plus pertinente à la crise des vocations. Nous le réaffirmons aujourd’hui : la meilleure réponse reste la reconnaissance du statut de l’élu local au moyen de dispositifs concrets, ainsi que la revalorisation du bloc communal. C’est pourquoi, afin de ne pas pénaliser les communes qui parviennent à constituer leur conseil municipal et de ne pas empêcher des conseillers municipaux de poursuivre leur engagement local, il semble de bon sens que la loi s’adapte aux spécificités communales

qui conduit, nous le savons tous, à une chasse aux élus, dans laquelle les maires et les adjoints sont souvent en première ligne, nous appelons à une réflexion plus large plus complète sur le mode de scrutin. La réduction de l’effectif légal dans les petites communes est un moyen de faciliter l’émergence de listes paritaires et donc égalitaires. Les avantages du scrutin de liste ont été mis en avant dans le rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales : ce scrutin favorise le bon fonctionnement des équipes municipales et garantit une parité plus efficace.

sont les garants du lien de proximité entre les administrés et les institutions. Ils veillent au bon fonctionnement des services publics, du moins ceux qu’il leur reste. Toutefois, nous devons aussi admettre que la multiplication des conseillers entraîne parfois, dans certaines communes, des difficultés à constituer les listes. Les conseils municipaux, lieux de démocratie, peuvent par ailleurs devenir des arènes où les débats s’éternisent et où l’administration locale souffre d’une lourdeur bureaucratique. La réduction du nombre de conseillers municipaux, associée au maintien du nombre d’adjoints, pourrait contribuer à dynamiser l’efficacité de ces instances décisionnelles. En resserrant le cercle des élus, nous faciliterions la coordination et la réactivité face aux défis auxquels nos communes sont confrontées. Avec un conseil plus restreint, la prise de décision serait plus rapide et fluide, ce qui permettrait de répondre de manière plus immédiate aux besoins des habitants. Cette proposition de loi favoriserait donc une gouvernance plus agile et plus moderne, adaptée aux réalités actuelles, quand les délais de réaction face aux urgences économiques, sociales ou environnementales sont de plus en plus courts. également un problème qui touche de nombreuses communes, à savoir le manque de participation démocratique des citoyens. Dans de nombreux territoires, nous observons une désaffection croissante des habitants pour la vie municipale : les taux de participation aux élections locales diminuent, les réunions publiques sont peu fréquentées et les initiatives participatives,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Alexis de Tocqueville disait : « C’est […] dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. » Qu’elle soit rurale ou urbaine, petite ou grande, la commune constitue la cellule de base, le fondement de la démocratie, et les élus municipaux, par leur engagement et leur abnégation, sont les maillons essentiels de la vitalité et du dynamisme de la démocratie locale.

Cette pénurie de candidats aux élections municipales peut porter atteinte à la démocratie locale. Ainsi, selon le rapport d’information de Mathieu Darnaud sur l’avenir de la commune et du maire en France, du maire en France, 106 communes ne disposaient d’aucun candidat lors du premier tour des élections municipales de 2020, soit une augmentation de 75 % par rapport aux élections de 2014. C’est beaucoup et c’est inquiétant.

La démocratie ne constitue pas un modèle figé. Elle doit accompagner les évolutions de nos territoires. Pour autant, si la réduction du nombre de conseillers municipaux répond à un réel problème auquel sont confrontés les maires de certaines petites communes,

Enfin, si cette initiative constitue un progrès, elle ne permettra pas à elle seule de traiter les causes de la crise de la démocratie locale que nous connaissons actuellement.

un choc de simplification est nécessaire, tous les élus nous le disent. Ils s’impatientent et nous sommes réellement heureux de vous savoir à nos côtés, pour à la fois prendre l’initiative et relayer nos préoccupations.

communes rurales, qui en ont besoin. Il faudra bien sûr – notre rapporteure l’a bien vu – neutraliser les effets de cette proposition de loi sur le nombre d’adjoints. se justifient non pas par le nombre de conseillers municipaux, mais par le nombre d’habitants, qui implique un certain niveau de service

puisqu’elles vivent sous le régime de la liste unique. Ce n’est pas un progrès de la démocratie. Veillons à l’avenir non pas à aggraver le déficit démocratique, mais au contraire à le combler.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, savez vous quel est le point commun entre Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Clemenceau, Francis Cabrel, Guy Roux et Stéphane Bern ?

n’est il pas paradoxal, tout en déplorant la baisse du nombre de conseillers municipaux actifs, de l’institutionnaliser et d’imposer ce que l’on regrette ?

du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes ne privera t elle pas notre pays de plusieurs dizaines de milliers de bonnes volontés si précieuses ?

de maintenir le nombre actuel de conseillers municipaux là où il n’y a pas de problème de recrutement et de le baisser là où il y en a ? Adaptons nous aux spécificités locales et municipales, selon la volonté municipale ! Nous savons volonté municipale ! Nous savons tous combien nous avons besoin des maires, des adjoints et des conseillers municipaux, de ces fantassins de la République qui sont toujours présents, toujours en première ligne. Plus ils sont nombreux, mieux c’est. Abondance de biens ne nuit jamais

En prévoyant de diminuer le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 500 habitants, ce texte répond à une forte attente des élus. Je me félicite que la commission soit allée plus loin en élargissant cette initiative aux communes de moins de 3 500 habitants tout en corrigeant les effets de bords du texte. Comme l’a souligné Mme la rapporteure, il est indispensable que cette baisse d’effectif n’emporte aucune conséquence sur le nombre d’adjoints. Traiter le symptôme est une chose, mais n’oublions pas de traiter les causes de ce désengagement, de ce désarroi local, équation insoluble qui fragilise l’engagement jusqu’à conduire, parfois, à la démission. À cela s’ajoutent les attentes nombreuses et légitimes de nos concitoyens et la complexité du millefeuille administratif. Les élus municipaux sont accablés, en première ligne face au désespoir et parfois à la violence, dans un contexte général d’« élu bashing ».

J’ai la conviction que certains ministres issus de notre assemblée sauront être force de proposition en la matière. Le Sénat répondra présent. Pour qu’une réforme puisse être applicable en 2026, il faudra rapidement se saisir du sujet. cette forte attente et sous réserve que le nombre d’adjoints soit conservé, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. La discussion

d’étendre l’assouplissement des règles numériques pour la composition des conseils municipaux des petites communes ayant des difficultés à composer un conseil municipal complet. Cette présomption de complétude, qui existe déjà dans les plus petites communes depuis l’adoption de la loi Engagement et proximité, doit être étendue aux communes de plus de 500 habitants et jusqu’à celles de 3 500 habitants, pour mieux tenir compte de la disparité démographique entre ces différentes communes. Le principe de complétude a l’avantage d’apporter de la souplesse à la logique des seuils sans pour autant pénaliser les communes ayant d’ores et déjà la capacité de réunir suffisamment d’élus.

Il conviendrait, en lieu et place d’une réduction du nombre de conseillers municipaux, de lutter contre le désengagement territorial de l’État dans les communes, en renforçant les ressources en ingénierie municipale pour aider les élus dans l’exercice de leur mandat et en prévoyant des ressources financières et fiscales suffisantes pour tenir compte de la complexification de leurs missions.

sans lien avec le nombre d’habitants. Une commune de 150 habitants pourrait avoir le même nombre de conseillers municipaux qu’une commune de 1 400 habitants, alors qu’elles sont de taille différente.

tandis que les communes de moins de 3 500 habitants pourraient choisir l’effectif de leur conseil municipal. Enfin, certains de ces amendements ont pour objet de supprimer la diminution des effectifs des conseils municipaux des communes comptant entre 500 et 3 500

demande du groupe Union Centriste, de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires, présentée par M. Philippe Folliot et plusieurs de ses collègues

contractuelle entre l’établissement et son client peut être rompue au nom de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – il s’agit, bien sûr, de sujets particulièrement sensibles.

que nous agirons en étroite collaboration. La proposition de loi de M. Folliot que nous examinons aujourd’hui vise à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires. À cette fin, elle entend garantir la transparence des motifs de clôture de comptes bancaires. Les banques seraient ainsi tenues de motiver, sur demande expresse du client, toute décision de résiliation unilatérale qu’elles prendraient à l’égard du compte de dépôt d’un client. et par ses collègues de la commission des finances, que je salue, ont permis de faire évoluer le texte, afin d’exonérer les établissements bancaires de cette obligation lorsque la divulgation du motif contreviendrait aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. De plus, il est désormais précisé que la banque dispose d’un délai de deux semaines pour répondre à la demande du client, sauf, bien sûr, si elle est autorisée à garder le silence. En tant que secrétaire d’État chargée de la consommation, je tiens à saluer l’initiative prise ici pour renforcer les droits des consommateurs

Comme vous le savez, les banques sont autorisées à clôturer un compte après avoir adressé une déclaration de soupçon au renseignement financier national. Mais, pour préserver l’efficacité de la lutte contre le blanchiment, la loi interdit aux banques de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur des opérations suspectes l’existence de cette déclaration. Cette confidentialité Cette confidentialité est essentielle à l’efficacité de notre renseignement financier : nous ne devons y toucher qu’avec une très grande prudence.

Depuis 1984, le législateur a d’ailleurs tenu à garantir l’accès aux moyens de paiement pour tous en gravant dans la loi le droit au compte, censé assurer l’accès à un service bancaire de base universel.

relation repose sur la contractualisation et sur un principe de réciprocité encadré par la loi, la force obligatoire du contrat et le code civil. Le client peut clôturer son compte bancaire sans préavis et sans justification.

Certes, l’usager, face à cette difficulté, n’est pas sans solution. En plus du préavis obligatoire de deux mois, il peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour l’ouverture d’un nouveau compte – le droit au compte. Mais de nombreux Français restent démunis pour engager cette démarche : il faut être informé de cette possibilité, connaître la Banque de France, savoir comment en faire la demande, quelle procédure suivre, etc. Cela peut être aisé pour une partie de nos concitoyens, mais, à coup sûr, plus complexe, voire insurmontable, pour certains d’entre eux. À cela s’ajoute le développement des démarches dématérialisées, qui multiplient les cas de non recours au droit.

Cette disposition utile lève la possibilité d’injonction contradictoire spécifique à la déclaration de soupçon. Vous l’aurez compris, l’évolution – légitime – prévue par ce texte va dans le bon sens,

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, sans compte bancaire, nulle activité sociale n’est possible : pas de versement de salaire, pas de versement de loyer, pas de pension de retraite.

L’obligation sociale de détenir un compte bancaire ne peut en effet s’accompagner d’une obligation de rentabilité. Sinon, c’est la double peine. Or, pour notre groupe, l’obligation sociale passe avant l’obligation de rendement – ce qui est un choix de société. Nous devons rompre avec le non droit bancaire, qui frappe les particuliers, mais aussi des entreprises. Mes chers collègues, nous avons examiné, sur la dernière session, cinq textes ayant trait aux comptes bancaires. Nous sommes face à un problème systémique

Nos concitoyennes et concitoyens sont confrontés aux commissions exorbitantes, aux ruptures abusives d’autorisation de découvert, au non respect des conventions de compte et aux refus d’exécution d’ordre. Ce système organisé a fait émerger des professionnels du litige bancaire

Cette organisation prospère sur la dissuasion des clients lésés, trop ignorants de leurs droits, trop pauvres pour se faire accompagner. Bref, c’est faire de l’argent sur le malheur des autres ! Tout cela a lieu dans un contexte où le résultat net des six principaux groupes bancaires progresse, en 2023, à, tout de même, 32,3 milliards d’euros. Pour la gestion des 2 179 milliards d’euros de dépôts des ménages, les banques facturent, selon la banque de France, « des commissions qui s’inscrivent à un niveau stable de 54,7 milliards d’euros et historiquement élevé ».

citoyens consommateurs. Perdre l’accès à un compte bancaire signifie souvent être privé de moyens de paiement, avec des conséquences directes sur la vie quotidienne. possible dans le contexte de bancarisation que nous connaissons : il faut donc y remédier. Deuxièmement, ce texte participe de la transparence que nous sommes en droit d’attendre du système bancaire.

Merci

En 2022, les établissements N26 et ING ont, en effet, été accusés de fermetures abusives sous couvert de lutte contre le blanchiment, aspect pris en compte, je le souligne, par le rapporteur. Les fermetures de comptes par Orange Bank, en 2024, avaient quant à elles touché 800 000 clients. Il est cependant difficile d’évaluer précisément le nombre de comptes clos abusivement chaque année. Pour les clients, les délais de remboursement des avoirs se révèlent longs et nombre d’entre eux se sont retrouvés sans accès à leurs fonds pendant des mois. Qui plus est, les justifications restent souvent vagues et les recours peu efficaces.

Actuellement, nos concitoyens peuvent contacter le médiateur bancaire ou rejoindre des collectifs d’usagers pour mener des actions communes. Cependant, ces démarches sont souvent longues et incertaines. La jurisprudence montre que les banques peuvent être tenues pour responsables en cas de fermeture abusive, mais il est nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice réel, ce qui n’est pas toujours évident. Selon la législation en vigueur, les établissements bancaires ont le droit de fermer un compte, mais doivent respecter un préavis de deux mois et en informer le client par écrit. La convention de compte, signée entre la banque et le client, régit ces procédures. L’apport principal de cette proposition de loi est l’obligation pour la banque de motiver la fermeture d’un compte.

Par ailleurs, le texte proposé ne prend pas en compte les différences de législation entre pays, ce qui soulève des difficultés pour les clients de néobanques dont les comptes sont domiciliés à l’étranger.

l’accès au système bancaire est un enjeu clé pour la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Sociale, d’abord, car sans compte en banque, l’intégration à la collectivité est difficile, sinon impossible. Se loger, travailler se nourrir

En milieu urbain ou périurbain, il est ainsi souvent possible de se rendre, à pied, dans plusieurs agences. En milieu rural, il n’est au contraire pas rare de devoir prendre sa voiture pour se rendre dans une seule d’entre Compte tenu de ces deux dimensions, on comprend que la fermeture de compte puisse être un facteur d’exclusion. C’est pourquoi je remercie nos collègues du groupe Union Centriste d’avoir inscrit ce texte à l’ordre du jour.

À la vérité, on ne le sait pas très bien… En 2019, une enquête menée par l’UFC Que Choisir estimait à 11 % la proportion de personnes déclarant avoir déjà fait l’objet d’une fermeture de compte par leur banque sans leur accord. Mais parmi ces fermetures, certaines étaient justifiées. La proposition de loi que nous examinons concerne les personnes dont le compte a été fermé sans leur accord, qui n’en comprennent pas la raison et qui ne peuvent ouvrir un compte dans une autre banque, soit en agence, soit en ligne.

c’était prendre le risque que rien ne change. En effet, vous connaissez tous le mot de Richelieu : « Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c’est autoriser la chose qu’on veut défendre. Le rapporteur, Marc Laménie, dont je tiens à saluer le travail et dont le groupe Les Indépendants soutiendra majoritairement la position, a réécrit, à juste titre, ce texte. Les banques seraient désormais obligées, lorsque le client en fait la demande, de motiver leur décision

la condition ajoutée pose tout de même une difficulté, car l’absence de réponse de la banque équivaut à faire peser un soupçon sur la personne concernée. Nous espérons donc que ce texte sera encore amélioré tout au long de son examen parlementaire.

je suis parti à l’étranger pour travailler et rejoindre ma famille, la banque m’a envoyé une lettre recommandée : “Nous n’avons plus convenance à maintenir la relation de compte que nous avons avec vous […]. Cette relation de compte prendra fin dans soixante jours.” Je n’ai pu obtenir une explication de la part de ma conseillère de clientèle. »

Ce compte bancaire leur permet en effet de recevoir la pension de retraite française, le remboursement de leurs soins et les loyers qu’ils tirent des biens dont ils sont propriétaires en France ; de payer leurs impôts en France, d’adhérer à une mutuelle ou de régler les études de leurs enfants ; ou, tout simplement, d’épargner. Quelles sont les raisons notifiées par les banques françaises aux Français de l’étranger pour ces fermetures ? Aucune, madame la secrétaire d’État ! Quelles sont les deux raisons invoquées par les collaborateurs bancaires ?

comme c’est le cas en Afrique de l’Ouest, au Moyen Orient ou en Amérique latine. La seconde est la réglementation extraterritoriale américaine du qui impose aux institutions françaises de déclarer aux autorités américaines les comptes détenus par des citoyens américains ou franco américains. Pour éviter de gérer des obligations complexes, les établissements français préfèrent clôturer les comptes de ces non résidents. Face à de telles régulations internationales, les banques, par prudence, surinterprètent des textes dont l’objectif initial n’était pas la fermeture de comptes bancaires. D’ailleurs, aucun des pays considérés comme étant sensibles ou à risque ne fait aujourd’hui l’objet d’une interdiction générale et absolue de transactions financières. Il n’y a donc aucune raison d’empêcher, par principe, des transactions par la fermeture de comptes bancaires. À ces Français dont la banque a subitement fermé le compte, l’on répond qu’ils peuvent exercer leur droit au compte, comme s’ils étaient des faillis ou des interdits bancaires.

peut, à son tour, clore le nouveau compte dans certaines situations. C’est notamment le cas lorsqu’elle prétend ne pas être en mesure de satisfaire aux obligations de vigilance, principales causes actuelles de fermeture des comptes des Français de l’étranger. Vous l’avez compris, la motivation d’une décision de fermeture d’un compte bancaire ou le rallongement du délai de préavis sont totalement inopérants pour résoudre le problème de la clôture des comptes bancaires des Français de l’étranger.

une situation inacceptable, estimant « anormal que les Françaises et les Français ici soient amenés à aller vers des banques étrangères parce qu’ils sont abandonnés par les banques françaises

mes chers collègues, le texte que nous examinons vise à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires. Notre groupe votera pour cette proposition de loi. Pourquoi ?

la législation en vigueur permet à une banque de résilier unilatéralement un compte bancaire sans avoir à se justifier sur les motifs de cette fermeture de compte. Autrement dit, si un client apprend que son compte bancaire fait l’objet d’une fermeture et qu’il souhaite en connaître les raisons, l’établissement peut, en toute légalité, ne pas indiquer les motivations de cette fermeture, laissant ainsi le client dans un flou sidérant. Est ce bien logique ? Non ! Une telle situation crée une incompréhension légitime et suscite peut être encore un peu plus de méfiance à l’égard d’un secteur déjà largement décrié… Ce texte rééquilibre la situation au bénéfice du client en lui permettant, s’il le demande, d’obtenir en toute transparence les raisons justifiant la fermeture de son compte en banque. Cette transparence éviterait des abus, à savoir les fermetures aléatoires ou injustifiées, raison pour laquelle nous sommes en faveur de l’adoption de cette proposition de loi. Toutefois, un certain nombre de zones d’ombre devront être éclaircies au cours de la navette parlementaire. Je pense, notamment, aux incertitudes juridiques, à commencer par celles qui concernent le droit communautaire. En effet, l’article 55 de la deuxième directive européenne sur les services de paiement, transposé dans le code monétaire et financier français, rappelle la faculté pour l’établissement de résiliation unilatérale du contrat cadre et la soumet à la seule condition de respecter un préavis de deux mois. La motivation de la résiliation n’est donc pas prévue en tant que telle par la directive, ce qui pose la question de l’éventuelle absence de conformité avec le droit de l’Union.

je souhaite également aborder une autre préoccupation : celle des conséquences de l’adoption de ce texte sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment. Si un client auteur de faits pouvant, par exemple, être qualifiés de blanchiment ou de financement du terrorisme découvre la décision de clôture de son compte bancaire, il pourrait dès lors considérer qu’il fait l’objet d’une enquête. Cela reviendrait donc ni plus ni moins à lui mettre la puce à l’oreille, lui laissant ainsi l’opportunité de procéder à la destruction de preuves utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité, et ce avant la fin de l’enquête. Je crains que l’amendement du rapporteur n’ait pas résolu ce problème dans la mesure où le refus de justification permettrait de raisonner, lui mettant une fois encore la puce à l’oreille. Face à de tels risques, j’ai donc déposé un amendement à ce sujet, en proposant une piste de réflexion. Malgré ces zones d’ombre, je pense néanmoins qu’il est nécessaire de ne pas laisser le droit en vigueur figé.

les Français établis hors de France sont les premières victimes, parfois tragiques, des fermetures abusives et arbitraires de comptes bancaires en France. Combien de fois n’ai je été confronté à ces retraités dont la seule source de revenus, leur petite retraite, devenait inaccessible ? Combien de fois n’ai je été sollicité par ces entrepreneurs français qui participent à notre commerce extérieur et qui voient leurs comptes bancaires brutalement et injustement fermés ? N’oublions pas non plus ceux que l’on appelle les Américains accidentels, particulièrement concernés. Ces fermetures abusives de comptes bancaires n’ont que trop duré. Il est enfin temps d’agir pour nos compatriotes établis hors de France. Depuis la loi bancaire du 24 janvier 1984, tout Français, qu’il réside dans l’Hexagone, dans les outre mer ou à l’étranger, a le droit de posséder un compte de dépôt dans une banque en France. C’est le droit au compte, prévu en particulier par l’article L. 312 1 du code monétaire et financier. Mais ce droit au compte est malmené. D’une part, pour des Français établis a à l’étranger, les décalages horaires, les délais postaux et la distance avec la France complexifient les procédures, surtout pour les naufragés du numérique. D’autre part, dans la plupart des cas, l’établissement bancaire désigné par la Banque de France n’offre que les seuls services bancaires de base, ce qui représente une détérioration du service rendu. En effet, de nombreuses banques ferment arbitrairement et abusivement les comptes de nos compatriotes établis à l’étranger après avoir notifié un préavis de deux mois. La lutte contre le terrorisme, la fraude et le blanchiment ne s’appliquent pas à ces Français à l’attitude irréprochable et exemplaire dont le seul crime serait de se battre pour le rayonnement de la France à l’étranger

ci fait référence à l’échange entre les autorités fiscales internationales, dans le but de réduire l’évasion fiscale mondiale et d’accroître la transparence fiscale. À cela s’ajoutent les recommandations du Groupe d’action financière (Gafi), qui définissent un cadre complet de mesures devant être mises mises en œuvre par les pays afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Concrètement, plutôt que de faire l’objet d’un examen au cas par cas, des Français de l’étranger voient injustement leur compte bancaire fermé, ce qui les place en grande difficulté. Nous soutenons donc cette proposition de loi, qui tend à protéger les Français de la fermeture abusive de leur compte bancaire en contraignant les établissements bancaires à se justifier. Or l’expérience a montré que les banques procédaient souvent sans discernement. Madame la secrétaire d’État, nous connaissons votre attention à la protection du consommateur et savons que nous pouvons compter sur vous, votre rigueur et votre ténacité. C’est pourquoi nous sommes d’accord avec vous pour que des travaux complémentaires d’analyse soient menés. À ce titre, nous saluons votre engagement à saisir le Comité consultatif du secteur financier de ce sujet, et nous serons attentifs à ses conclusions. La lutte contre le blanchiment est évidemment une dimension essentielle, à laquelle nous sommes attentifs. Au delà de cette proposition de loi, formons ici le vœu que la Fédération bancaire française (FBF) et le gouverneur de la Banque de France entendent notre appel à plus de justice pour les Français de l’étranger. les Français de l’étranger. Ceux d’entre eux qui détiennent un compte bancaire en France ne sont ni des fraudeurs, ni des criminels, ni des exilés fiscaux, mais ils ont besoin d’un tel compte pour de multiples raisons : régler leurs impôts, percevoir une retraite, régler des frais de scolarité, acquitter une pension alimentaire, etc. Nous sommes ici leurs avocats face aux abus bancaires qui les frappent.

largement dématérialisés l’espace client ou par courriel. Enfin, avec une offre bancaire large et concurrentielle d’établissements en ligne, le marché français est adapté pour répondre dans des délais courts à une ouverture de compte, même opérée

En parlant de fermetures abusives de comptes bancaires, on minimise la réglementation déjà existante, qui impose un préavis de deux mois et consacre le droit au compte. Les banques n’ont tout simplement pas d’intérêt à fermer un compte. En plus d’alourdir les procédures avec une obligation purement formelle, on stigmatise des employés de tout un secteur qui sont largement présents dans nos territoires et s’imposent comme des acteurs du développement économique local. Ce sont bien les employés chargés d’accueil ou de clientèle et les directeurs d’agence qui seront directement exposés, dès lors qu’ils sont déchirés entre plusieurs règles contradictoires.

inenvisageable pour un conseiller, s’il fallait le préciser, d’indiquer à son client que son compte est fermé pour soupçon de financement du terrorisme. L’amendement adopté en commission, résultant du travail constructif de mon collègue Marc Laménie, va dans le bon sens puisqu’il tend à poser une exception lorsque la motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Toutefois, il ne règle qu’une partie du problème. Si le conseiller ne justifie pas au client la fermeture de son compte, ce dernier pourra aisément en déduire qu’on le soupçonne et ainsi prendre les dispositions nécessaires. On imagine bien la situation délicate dans laquelle se retrouverait un conseiller face à un tel client. En plus d’affaiblir l’action commune des autorités, des établissements bancaires et de Tracfin dans la lutte contre le financement du terrorisme

Si l’obligation pour les banques de justifier la clôture d’un compte bancaire était systématisée, même en l’absence de demande du client, cela contribuerait à aggraver le conflit de normes avec le principe de confidentialité de la déclaration

soit contrevenir à la loi en présentant des motivations inexactes pour préserver la confidentialité de sa déclaration de soupçon. Nous retrouvons donc ici les

et la poursuite ou non de la relation d’affaires, dont la décision revient à la banque concernée. Le fait pour une banque de maintenir un compte ouvert, alors qu’elle sait que l’activité du compte est liée à des infractions pénales, est susceptible de rendre celle ci, avec ses dirigeants, complice d’un crime ou d’un délit